J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.

à répondre aux difficultés de ces professionnels et à prendre en compte les charges pesant sur les directeurs d'établissement scolaire. Tout d'abord, de même que nous nous opposons au recrutement direct des enseignants, il nous semble essentiel de garder un cadre national des affectations en matière d'AESH. En effet, cette pratique participe à la dynamique visant à appliquer dans le service public, par ailleurs régalien, les mêmes logiques managériales et gestionnaires que dans le secteur privé. La situation actuelle tend à faire des écoles et des établissements du secondaire des unités totalement indépendantes, et non des maillons du système plus global que devrait être l'éducation nationale. Ensuite, un tel recrutement met les AESH directement sous la responsabilité et les ordres des directeurs d'établissement. De fait, cela conduit à empêcher une uniformisation de leurs conditions de travail, notamment en matière d'accès aux réunions pédagogiques et de tâches dévolues à ces accompagnants. Comme le signalent depuis plusieurs années les professionnels du secteur, certaines académies et certains établissements ont tendance à user de leur pouvoir hiérarchique pour imposer aux AESH des tâches qui ne devraient pas les concerner. Je pense notamment à la pratique d'actes médicaux ou paramédicaux, à l'accompagnement sur du temps périscolaire et extrascolaire, voire à la transformation des AESH en véritables assistants des enseignants. En parallèle, selon leur employeur, ces professionnels peuvent se voir autoriser ou refuser l'accès à des réunions pourtant essentielles à leur activité. Enfin, il faut bien le rappeler, les directeurs d'établissement ont déjà suffisamment de tâches pour ne pas avoir à gérer en plus le recrutement des AESH. C'est d'autant plus vrai que l'argument parfois avancé par le ministère laisse dubitatif. Ainsi, les directions d'établissement seraient les plus à même d'évaluer les besoins d'accompagnement des élèves de leur établissement. Sauf à considérer que les directeurs sont tous des experts de la sensibilisation et de l'accompagnement du handicap, on voit mal comment ces derniers pourraient être plus qualifiés et compétents que les spécialistes des maisons

permettrait d'établir une circulaire de cadrage aux rectorats, harmonisant l'ensemble des conditions de travail des AESH, notamment s'agissant du temps de travail. part, d'après les informations qui nous sont remontées, le recrutement par les collectivités, pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement, n'apparaît pas satisfaisant pour le développement de l'autonomie des élèves handicapés en contact avec le même AESH pendant le temps scolaire et en dehors pour d'autres activités. Monsieur le ministre, vous avez avancé des arguments qui n'allaient pas en ce sens. Mais

est à Mme Laure Darcos. Les AESH sont recrutés parmi les candidats titulaires du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, diplôme de niveau V, dont la création est relativement récente, voire sans condition de diplôme dès lors qu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'au moins neuf mois dans les domaines de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, des élèves en situation de handicap ou des étudiants en situation de handicap. Ils sont membres à part entière de l'équipe éducative. Comme le souligne le rapporteur, le nombre d'élèves scolarisés en situation de handicap a presque doublé entre 2004 et 2017, pour atteindre 391 000. Cette augmentation, due, entre autres, à l'élargissement du champ de la définition du handicap à des publics nouveaux, à un meilleur repérage des troubles, à des changements dans l'acceptation d'enfants handicapés qui peuvent être pris en charge ou encore à la progression de la poursuite d'études en milieu ordinaire dans le second degré, est intégralement réalisée en milieu ordinaire. Alors que la demande de suivi individuel ou mutualisé des élèves handicapés explose et que le milieu scolaire ordinaire accueille une plus grande diversité de handicaps, le besoin de formations adaptées se révèle particulièrement aigu, de l'avis même des accompagnants, qui jugent indispensable un renforcement de leur professionnalisation. Le présent amendement tend

d'AESH référents, que nous créons dans le projet de loi, les perspectives d'évolution professionnelle restent entières. Je considère votre amendement comme un amendement d'appel. Je vous suggère donc de le retirer, faute de quoi je serais obligé d'émettre un avis défavorable.

n° 91 rectifié. Certes, je partage l'esprit de ce qui est proposé. Nous allons en effet faire le maximum pour ouvrir des perspectives de carrière aux AESH. C'est d'ailleurs l'un des objets du dialogue social qui a lieu en ce moment même

Le rôle du référent AESH départemental est essentiel pour ses collègues, notamment pour ceux qui sont inexpérimentés. Les référents bénéficient d'une décharge pour accueillir et conseiller les nouveaux AESH.

il sera impossible pour un seul AESH de réaliser sa mission de maillage départemental de manière satisfaisante en devant sillonner des centaines de kilomètres dans une même journée, souvent en l'absence transports rapides, voire de transports tout court. tout court. Dans les départements ruraux comme le mien- le Lot -, il n'y a pas de transports en commun. Les référents devront forcément utiliser leur voiture et emprunter des routes départementales,

est à M. Claude Malhuret. Le code de l'éducation prévoit que les élèves intellectuellement précoces bénéficient d'aménagements particuliers, afin de favoriser leur intégration et leur réussite scolaire. Cet amendement vise à favoriser la réussite scolaire des enfants à haut potentiel, en précisant que l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences s'accompagne de mesures permettant à la communauté éducative d'adapter la scolarité des élèves intellectuelles précoces à leurs besoins éducatifs particuliers. Comme le mentionne la « mission flash » sur la prise en charge à l'école de la précocité et des troubles associés, il s'agit de généraliser les initiatives vertueuses prises par certains établissements scolaires pour adapter la scolarité des enfants précoces en difficulté. Ces mesures d'inclusion scolaire constituent une solution de substitution à la déscolarisation et un levier d'action contre l'échec scolaire, échec qui concerne encore un enfant surdoué sur trois.

à compter de la publication de la présente loi, à faire un état des lieux des besoins en personnels accompagnant les élèves en situation de handicap. Il faudra également envisager les évolutions possibles de leur statut et de leur formation.

amendements tendent au même objet pour différents types d'établissements dépendant de niveaux de collectivités différents. Le texte prévoit que tout projet de réhabilitation et de construction d'un établissement entraîne pour la collectivité concernée la prise en compte des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement. Nous avons évoqué, monsieur le ministre, la coopération

des établissements médico-sociaux et des centres d'action médico-sociale précoce. Il s'agit d'une demande des personnels qui oeuvrent sur le terrain au plus près des élèves. De ce fait, ils auront certainement des remarques pertinentes à transmettre sur l'adéquation des projets de travaux avec la situation

au conseil municipal, départemental ou régional de tenir compte des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.

de plus en plus nombreuses constituent des injonctions quelque peu contradictoires et mettent les élus en grande difficulté. Toutefois, la commission est aussi attachée au respect des prérogatives des commissions départementales d'élus locaux, par exemple la DETR, à qui il revient de décider des catégories d'opérations prioritaires. J'émets donc un avis défavorable

Il y a quelques années, on a même envisagé de le démolir pour le reconstruire. Les malfaçons sont nombreuses, ce qui entraîne beaucoup de réparations, mais les subventions de fonctionnement sont totalement insuffisantes. L'an L'an dernier, un plafond s'est effondré, heureusement en dehors des horaires de cours, sans quoi des élèves auraient été tués ou blessés, et c'eût été un carnage ! La réhabilitation des bâtiments d'enseignement à Wallis et à Futuna devra avoir lieu d'urgence, et en tenant compte des nouvelles normes de sécurité. Il y va de la sécurité et de la vie des élèves et des enseignants.

du Gouvernement ? Dans le cadre des opérations de construction ou de réhabilitation des établissements dont l'État à la charge à Wallis et à Futuna, les recommandations pour une école inclusive, émises par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement ont évidemment vocation à être prises en compte. Toutefois, dans une logique de cohérence avec les autres dispositions relatives à Wallis et à Futuna, il paraît préférable de traiter ce point dans le cadre des dispositions prévues à l'article 22 du projet de loi. Pour cette raison, j'émets un avis défavorable

Renouer la confiance avec les familles d'élèves handicapés nécessite de faciliter les parcours scolaires et de garantir aux parents la reconnaissance et la prise en compte des besoins spécifiques de leurs enfants, ainsi que la mobilisation plus rapide de réponses adaptées. La réussite des parcours scolaires des élèves handicapés implique une coopération plus étroite de l'ensemble des professionnels de l'éducation nationale et du secteur médico-social, avec comme objectif une école toujours plus inclusive. Il s'agit, concrètement, de renforcer la présence et l'intervention des équipes médico-sociales au sein des établissements scolaires, en complémentarité des dispositifs d'inclusion scolaire existants. L'amendement tend à conforter le cadre de la coopération entre les deux secteurs, afin de permettre celle-ci en toutes circonstances, y compris en anticipation d'une éventuelle décision de la MDPH. Il vise à ouvrir la possibilité qu'un enfant handicapé et/ou l'équipe l'équipe pédagogique bénéficient d'un appui apporté par une équipe médico-sociale déjà présente dans l'école, une équipe mobile ou un pôle de compétences et de prestations externalisées. En cela, il tend à sécuriser, donc à favoriser la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés.

afin que les élèves sportifs scolarisés dans les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger bénéficient également des aménagements horaires et d'une scolarité adaptée.

Les quelques élèves des établissements de l'AEFE concernés par le sport de haut niveau bénéficient déjà de possibilités d'aménagement de leurs horaires. L'AEFE nous l'a confirmé

La loi pour la modernisation de notre système de santé a permis l'organisation des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, les ITEP, en « dispositifs intégrés », destinés, dans le cadre de la stratégie de transformation de l'offre médico-sociale, à favoriser des modalités d'accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qu'ils accueillent, en lien avec leurs parcours scolaires. L'évaluation de ce dispositif a conclu à l'utilité de l'élargir à l'ensemble des établissements et services médico-sociaux accompagnant des jeunes en situation de handicap. Le fonctionnement en dispositif intégré est en effet un réel moyen de permettre une meilleure fluidité des parcours et, ainsi, d'améliorer l'inclusion scolaire, en assurant la mobilisation plus rapide de réponses adaptées. Ce dispositif permet en effet de renforcer la scolarisation dans l'école ordinaire de façon sécurisée pour les enfants concernés, puisque l'accompagnement peut être adapté et reconfiguré rapidement au fil du temps. Cet amendement tend à élargir à l'ensemble des établissements et services médico-sociaux accompagnant les jeunes en situation de handicap la possibilité de s'organiser en « dispositif intégré

Monsieur le ministre, Les dispositifs intégrés permettent aux jeunes des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, les ITEP, de bénéficier d'une réorientation vers le milieu ordinaire, sans passer par une nouvelle saisine de la CDAPH. L'amendement vise à étendre les dispositifs intégrés à d'autres établissements médico-sociaux.

La qualité des coopérations entre les établissements et les différentes institutions qui encadrent et accompagnent la mise en oeuvre de ces politiques est fondamentale. C'est cohérent avec ce que nous disons depuis le début sur la notion de réseau, sur la fluidité et sur le travail en équipe. objectif partagé est en effet que les élèves soient réellement bénéficiaires de cette évolution et que les enseignants et les cadres disposent d'un appui solide et constant de la part des personnels spécialisés des établissements médico-sociaux. Il nous faudra ensuite préparer le décret et les conventions permettant de structurer l'accomplissement de cet objectif.

L'article 6 institue le cadre législatif applicable aux établissements publics locaux d'enseignement international. Ces derniers vont pouvoir s'implanter sur tout le territoire en fonction de la volonté des collectivités territoriales, prenant exemple sur l'école européenne de Strasbourg, qui est une référence et un succès. Ces établissements seront constitués de classes de premier et de second degré, qui dispenseront des enseignements en langue française et en langue étrangère. Ils prépareront à l'option internationale du brevet, au bac et au bac européen. Ils seront non seulement un levier indéniable d'attractivité à l'international, mais aussi un vecteur de rayonnement local. Les EPLEI participeront ainsi à l'objectif d'enrichissement de l'offre de formation et d'adaptation des structures administratives locales, tel qu'il est visé par le projet de loi pour une école de la confiance. De plus, l'admission des élèves se fera après la simple vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dans la langue étrangère pour laquelle ils se portent candidats, le tout dans des conditions adaptées à leur âge. Ces établissements n'ont pas vocation à devenir élitistes. Ils donneront ainsi à nos élèves toutes les chances d'avoir un acquis linguistique et culturel important, qui leur favorisera, j'en suis convaincu, la meilleure insertion professionnelle en France ou à l'international. à la lecture de l'arrêté du 18 janvier 2019 fixant la liste des sections internationales, il apparaît que les États limitrophes des départements d'outre-mer pouvant bénéficier de telles conventions sont quasi inexistants. Aussi, pour une meilleure insertion de ces territoires dans leur environnement géographique, je proposerai, un amendement, une demande de rapport d'évaluation de cette mesure dans les deux ans, afin de

Lepage, sur l'article. Nous abordons dans cet article 6 la création des établissements publics locaux d'enseignement international, ou EPLEI. En tant que sénatrice représentant les Français établis hors de France, attachée au plurilinguisme, je ne peux qu'approuver la création d'écoles qui promeuvent des enseignements en langue vivante étrangère. Nous ne pouvons en effet que nous réjouir de voir de futurs élèves devenir parfaitement bilingues, voire trilingues à la sortie de leurs études secondaires, comme c'est souvent le cas dans les établissements du réseau d'enseignement français à l'étranger. De plus, il convient que les enfants des salariés des organisations européennes ou internationales, à qui ces EPLEI s'adressent en priorité, puissent bénéficier d'un enseignement dans leur langue maternelle, en allemand, en anglais ou dans une autre langue. C'est pourquoi, au vu de ce contexte, le fait que l'admission des élèves soit soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dans la langue de la section pour laquelle ils sont candidats ne me semble pas poser de difficultés majeures, même si un test peut se révéler inutilement stressant pour les plus jeunes et si les enfants de 3 ans peuvent apprendre une langue très rapidement. Par ailleurs, si notre pays souhaite à l'avenir accueillir ces organisations internationales, la création de ces établissements est un préalable nécessaire. Cependant, je m'interroge sur le fait que ces futurs EPLEI, qui relèvent de la tutelle conjointe du ministère de l'éducation nationale et du Conseil des écoles européennes, prépareront soit à l'option internationale du diplôme du diplôme national du brevet et du baccalauréat, soit au baccalauréat européen. Or ce sont des programmes différents, des pratiques différentes, qui ne s'adressent pas au même public et n'ont pas les mêmes objectifs. L'instauration de ces établissements ne doit surtout pas nous faire oublier, mes chers collègues, l'immense défi que représente l'enseignement des langues étrangères au sein de notre pays. Chaque élève devrait pouvoir maîtriser une langue étrangère au moins à la fin de ses études secondaires, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Monsieur le ministre, au côté de ces nouveaux établissements, il est indispensable de développer, sur l'ensemble du territoire, des sections internationales, qui permettent d'intégrer, au sein du système français, un enseignement ouvert sur le monde. Ce n'est que par cette politique ambitieuse que nous parviendrons définitivement à mettre un terme à l'échec relatif de l'enseignement des langues vivantes en France.

me semble particulièrement adaptée à la situation des départements français d'Amérique, qui, comme vous le savez, sont entourés de territoires anglophones et hispanophones. J'irai plus loin : je reste persuadé que l'enseignement bilingue doit être la norme dans ces collectivités. Ainsi, une réflexion spécifique à ces territoires aurait pu éviter deux écueils, qui rendront très peu probable la création d'EPLEI dans les outre-mer : le premier est financier, et le second relatif à l'absence de prise en compte de l'environnement linguistique régional des outre-mer. Financièrement, les collectivités ultramarines auront des difficultés à faire face aux obligations qui leur incomberaient avec la création d'un nouvel établissement. Sur le principe, à la faveur de la création des EPLEI, une réflexion de fond aurait pu être conduite sur l'opportunité de différencier véritablement les enseignements en outre-mer. De fait, en 2011, à la suite d'une mission sur le tourisme en Guadeloupe et en Martinique, j'avais constaté la nécessité d'ouvrir les Antilles à d'autres marchés et à d'autres cultures, pour favoriser notamment la fin d'une vision « coloniale » du tourisme qu'une orientation longtemps exclusivement tournée vers la métropole a pu alimenter. alimenter. La barrière de la langue a sans doute aussi été à l'origine de cette orientation et de son alimentation. Aussi, pour doper l'activité et modifier la culture touristique, le bilinguisme me semble devoir être l'objectif à atteindre à l'issue du second cycle, ce qui favoriserait de surcroît

et aux engagements que vous pourrez prendre au nom du Gouvernement- ils détermineront mon vote sur cet amendement. La parole est à M. Guillaume Gontard, sur l'article. Monsieur le président, je reprends une intervention de ma collègue Esther Benbassa, La création d'établissements publics locaux d'enseignement international prévue à l'article 6 participera sans nul doute au renforcement de l'attractivité du système éducatif français et peut permettre, à terme, d'adapter l'offre scolaire des territoires. Cependant, la mise en oeuvre de ce dispositif nous pose problème. Ainsi, nous regrettons les modalités d'admission des élèves, calquées sur celles qui sont en vigueur à l'école européenne de Strasbourg, à savoir une sélection drastique fondée sur le multilinguisme de l'élève dans une langue européenne. Or, nous le savons, le multilinguisme est bien souvent l'apanage des familles les plus aisées, celles dont les enfants reçoivent très tôt un apprentissage des langues étrangères. La réalité est tout autre : selon une étude réalisée par Education First, la France se trouverait au 22 rang sur 26 pays européens en ce qui concerne les langues étrangères après la Roumanie et la Bosnie-Herzégovine. La France, pays mondialisé, devrait développer des écoles internationales, mais, en pleine crise sociale, il serait parfaitement regrettable de ne pas pouvoir intégrer dans ce nouveau cursus des élèves issus des diverses strates de la société. Pourquoi exclure la mixité sociale dans les formations d'excellence, en instaurant des prérequis dès le plus jeune âge ? Nous sommes bien loin du principe d'égalité de l'école républicaine ... Un tel élitisme institutionnalisé risque d'accroître l'inégalité des chances entre les élèves, et ainsi perpétuer l'injustice au sein de notre société.

En premier lieu, les EPLEI pourront préparer, au sein d'une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat et du diplôme ou de la certification permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans un État étranger en application d'accords passés avec cet État. Je crois que cette mesure lève l'une des objections que j'ai entendues. La rédaction actuelle, qui évoque uniquement le baccalauréat général, ne permet pas d'inclure les filières technologiques qui entrent pourtant dans le dispositif actuel des sections binationales. Il est donc proposé de supprimer la référence au caractère général du baccalauréat. En second lieu, la diversité de l'offre de formation d'un certain nombre d'établissements qui souhaitent accéder au statut d'EPLEI justifiait d'offrir à ce type d'établissement la possibilité de dispenser des formations préparant au diplôme de droit commun- brevet des collèges ou baccalauréat général, technologique ou professionnel. Afin de conserver la spécificité des futurs EPLEI, ces formations ne pourront pas être suivies par plus d'un quart de l'ensemble des effectifs de l'établissement. C'est le sens du nouvel alinéa proposé. Enfin, cette ouverture des EPLEI à des formations préparant aux diplômes de droit commun implique d'ajuster les dispositions relatives à l'admission des élèves, en limitant les tests d'admission aux seuls élèves souhaitant accéder aux formations linguistiques spécifiques. De plus, il est préférable de faire référence à la langue de la section, plutôt qu'à la langue étrangère, puisqu'il peut exister, au sein des écoles européennes, une section francophone. Ces modifications ajoutent de nouvelles garanties en matière de mixité sociale au sein des EPLEI, en leur permettant de préparer une partie des élèves au brevet des collèges et au baccalauréat général, technologique et professionnel. Cela s'accompagnera aussi de mesures pratiques afin que, de façon volontariste, toutes les classes sociales soient

de cette ségrégation économique et spatiale, la seule solution, monsieur le ministre, c'est que l'État investisse beaucoup plus dans les territoires qui en ont besoin. Je donnerai un autre exemple. Je suis conseiller départemental

que des jeunes qui viennent d'un peu plus loin, parce qu'ils ont un intérêt particulier à suivre la section arable, allemande, portugaise, etc. Ce type de lycée existe, et c'est ce qu'il faut développer. Je ne me suis peut-être pas exprimé très clairement par rapport par rapport à l'établissement de Strasbourg. Au départ, j'étais partie sur l'idée de l'école européenne. Je connais ce modèle d'établissement pour en avoir

accueillir des enfants du secteur, mais aussi développer les sections internationales. Nous avons besoin d'étendre l'enseignement des langues au-delà de deux heures par semaine. Nos enfants doivent être en mesure de mener une vraie discussion et de conduire un vrai travail dans des langues étrangères.

aux zones REP et REP+. Il s'agit vraiment, monsieur le ministre, de vous prendre au mot et de préciser dans la loi que nous voulons ensemble faire de ce nouveau dispositif un véritable outil d'égalité des chances. Je comprends les intentions des auteurs de l'amendement. Toutefois, l'initiative de créer un EPLEI repose exclusivement sur les collectivités territoriales concernées.

je rejoins le rapporteur pour dire que l'on ne doit pas introduire une rigidité supplémentaire. On doit respecter les choix des collectivités locales, sachant que l'éducation nationale aura vocation à encourager les implantations volontaristes dans certains territoires qui pourront ainsi se requalifier. Le Gouvernement

On peut imaginer que l'adoption de notre amendement permettrait au ministre d'engager une concertation avec les associations d'élus pour examiner comment, sur plusieurs années, installer et développer ces établissements que vous ne cessez de nous vanter au nom de la mixité sociale. Toutefois, quand il faut passer aux actes,

La création des établissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux, les EPLESF, ou des établissements publics locaux d'enseignement international, les EPLEI, modifie profondément les équilibres entre le premier et le second cycle. Cette modification porte atteinte à la relation de proximité, nécessaire et précieuse, entre les familles et le directeur d'école, le directeur d'école et son équipe éducative, le directeur d'école et la commune.

La composante « école » de l'établissement demeurera dirigée par un directeur d'école. Toutefois, pour que l'établissement fonctionne bien, il convient, dans le cadre des EPLEI, que le chef d'établissement ait bien autorité sur l'ensemble de l'établissement, comme c'est d'ailleurs le cas dans les

que beaucoup de pays limitrophes des départements d'outre-mer n'apparaissent pas dans la liste fixée par l'arrêté du 18 janvier 2019. Rappelons que les EPLEI préparent soit à l'option internationale du diplôme national du brevet et à l'option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen. Ces établissements seront créés par arrêté du représentant de l'État dans le département, sur proposition conjointe des collectivités territoriales. Il s'ensuivra une convention. En conséquence, on peut s'interroger sur le financement des établissements publics locaux d'enseignement international, compte tenu de la fragilité financière des collectivités territoriales des départements d'outre-mer. N'aurait-on pas plus de chances d'avoir des EPLEI en Île-de-France qu'en Martinique, en Guyane ou à Mayotte Dans cette logique, un rapport, après deux ans d'application de la présente loi, devrait nous permettre d'avoir une bonne visibilité sur la création et la gestion des EPLEI dans les outre-mer. Mes chers collègues, à titre exceptionnel, je vous encourage à adopter cet

duquel, dans les EPLEI formant un unique établissement, le conseil d'administration est censé exercer les compétences d'un conseil d'administration normal.

territoriale dans les outre-mer. Je l'ai dit dès le début, la problématique est intéressante. Elle correspond à une nécessité absolue pour le développement des outre-mer dans leur espace régional, en particulier pour le développement de l'activité touristique, qui reste,

présenter l'amendement n° 67 rectifié . Les langues et cultures régionales constituent un patrimoine national et ne peuvent donc être traitées comme les langues étrangères. Leur apprentissage donne lieu à des activités qui contribuent directement à l'acquisition du socle commun, notamment pour la découverte du milieu.

l'organisation concrète de l'enseignement, on se retrouve avec une concurrence entre les langues régionales et les langues étrangères dans l'enseignement. Je n'ai pas besoin d'aller prendre l'exemple de ma grand-mère ; le mien

qu'il aurait défendu dans des épisodes précédents les langues régionales et que je ne serais pas allé dans le même sens

comme étant tous dans le même bateau, le bateau « France », avec une langue qui est le français, consacrée par la Constitution, et des langues régionales, qui participent de la vitalité générale du pays.

en faveur des langues régionales. Je voudrais citer un exemple, qui a été trop peu souligné à mes yeux : dans le cadre de la réforme du lycée, l'un des enseignements de spécialité peut être l'enseignement d'une langue régionale, ce qui est

du Conseil constitutionnel est très claire à cet égard, puisque celui-ci a jugé à plusieurs reprises que l'enseignement des langues régionales, s'il pouvait être encouragé, ne saurait avoir un caractère obligatoire ni pour les élèves ni pour les professeurs. Il y a eu plusieurs décisions en

de ceux qui se sont mobilisés depuis des décennies sur les langues régionales et qui craignent qu'une victoire symbolique sur le socle ne se trouve remise en cause dans l'organisation concrète. D'où l'importance de cet amendement. Je le regrette, monsieur le ministre, mais ce n'était pas le sens de votre réponse.

que vous n'ayez pas, pour les langues régionales, pris les dispositions qui valent pour les sections internationales ou les sections européennes. Il y a là incontestablement un vrai problème et une véritable inquiétude, que Ronan Dantec

Le magnifique tableau que le ministère a publié pour les sections internationales et les sections européennes aurait pu aussi être publié pour les sections bilingues en langues régionales ; nous n'aurions pas alors les inquiétudes que Ronan Dantec a fort justement développées.

Antilles, nous sommes élevés dans une langue qui n'est pas exactement le français. Nous vivons avec le français. Nos petits traduisent bien souvent la langue créole quand ils parlent français. Éviter

Les choses sont donc très claires. Pour ma part, je suis évidemment partisan de donner un statut, et le plus haut possible, aux langues régionales, parce qu'il y va de la construction, je dirais même de la reconstruction

je vais lire à haute voix : « Dans les régions et territoires concernés, l'apprentissage de la langue et de la culture régionales est intégré au socle commun de connaissances, de compétences et de culture des élèves qui suivent cet enseignement. À ce titre, l'apprentissage de la langue et de la culture régionales doit être organisé de telle sorte que les élèves puissent le suivre sans être contraints de choisir entre cet enseignement et celui des autres domaines du socle.

Le scrutin est ouvert.

tel qu'il est. Mes chers collègues, il est minuit passé. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à minuit trente, afin de poursuivre l'examen de ce texte. Il n'y a pas d'observation

afin de permettre d'atteindre une véritable compétence bilingue des élèves, l'objectif de pleine maîtrise de la langue française étant assuré conformément à l'article L121-3 du code de l'éducation, qui est ici rappelé. Ce soutien particulier à la langue régionale, dans des contextes de diglossie au préjudice de la langue régionale, loin de nuire à la langue française, la renforce, au contraire. Le bilinguisme contribue au développement de hautes compétences dans les deux langues, notamment métalinguistiques, et favorise l'acquisition d'autres langues. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs validé ces différentes formes d'enseignement bilingue par sa décision 99-412 du 15 juin 1999, estimant qu'aucune des 39 dispositions de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires signées par la France le 7 mai 1999, y compris l'enseignement en immersion, n'était contraire à la Constitution.

nous avons eu, en effet, un échange un peu tendu avec Mme Gourault lors du débat sur la collectivité européenne d'Alsace -existe à l'école maternelle publique, dans le cadre de l'expérimentation.

je ne connais pas, moi- mais vous m'en présenterez peut-être -, d'enfants qui soient passés par des systèmes immersifs de langues régionales et qui ne parlent pas le français ! Je rappelle même que, voilà quelques années, le lauréat du concours général en français était un élève de l'école Diwan. Ce que vous dites n'est pas la réalité.

Monsieur le rapporteur, vous avez bien dit que l'aspect immersion se situait plutôt dans le cadre de l'expérimentation. Aujourd'hui, les écoles Diwan, mais aussi les écoles Calandreta en Occitanie, font de l'immersion

Le scrutin est ouvert.

Depuis 1996, les recommandations de La Haye concernant les droits des minorités nationales à l'éducation préconisent l'emploi de la langue maternelle de l'enfant comme vecteur idéal de l'enseignement au niveau de l'école primaire. En Guyane, dans la plupart des villages riverains du Maroni, le fleuve frontière avec le Suriname, et de l'Oyapock, le fleuve frontière avec le Brésil, ainsi que sur le littoral, qu'ils soient amérindiens ou bushinengués, c'est-à-dire descendants de noirs marrons, nos enfants n'ont pas le français pour langue maternelle. La reconnaissance de l'identité de ces peuples nous impose le respect et la défense de la spécificité de chacune de leurs langues, qui sont d'ailleurs reconnues comme langues de France. Dans cet esprit, la loi pour la refondation de l'école de la République a admis la possibilité du recours à ces langues pour l'acquisition du socle commun de connaissances. L'académie de Guyane a ainsi conforté la place de nos langues et de nos cultures, avec l'ambition forte de se doter, à moyen terme, de plusieurs écoles primaires bilingues.

Nous savons bien que l'échec scolaire de nos enfants est dû, en grande partie, à leurs difficultés à entrer dans les processus d'apprentissage de la lecture et de l'écriture du français. C'est pourquoi, parallèlement à l'abaissement à 3 ans de l'instruction obligatoire, il est indispensable de renforcer la prise en compte du plurilinguisme, pour garantir à ces enfants les mêmes chances de réussite. Pour atteindre cet objectif, les intervenants en langue maternelle sont précieux, mais ils ne suffisent Il faut également former les enseignants aux enjeux du plurilinguisme et accorder à ce dernier une place toute particulière dans le système éducatif des territoires ultramarins. Il serait temps de faire de cette richesse linguistique ce qu'elle est : un atout inestimable pour les jeunes.